Cet amendement porte sur le délai de rétractation précédemment discuté. Le droit à l'image et à l'identification est un sujet sensible et délicat. Or la formulation initiale prévoyait que les personnes enregistrées puissent rétracter leur consentement dans un délai de quinze jours à dater de l'audience. Au vu des circonstances d'un procès, qu'il soit civil ou pénal, une des parties au procès, dans la difficulté de la situation

de prendre une décision en pleine connaissance des éléments qui seront diffusés. Tel est l'objet de cet amendement.

L'article 1 apporte plusieurs garanties en matière d'enregistrement des audiences, en soumettant notamment à un accord écrit l'enregistrement des audiences qui ne sont pas publiques ou portent sur des litiges auxquels un mineur ou un majeur protégé Est également soumise à un accord écrit la diffusion de l'image et des autres éléments d'identification des personnes enregistrées. Afin de renforcer ces garanties, nos rapporteurs ont utilement inscrit dans l'article 1 le fait que cet accord écrit ne peut faire l'objet d'aucune contrepartie. garantie soit effective, le présent amendement tend à l'assortir d'une sanction, en lui appliquant le quantum d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, prévu par ailleurs par l'article, lorsqu'une diffusion méconnaît les conditions qu'il pose. Il apparaît en effet indispensable, pour que cette garantie supplémentaire soit effective, d'assortir sa méconnaissance de sanctions. Je pense que notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie n'aurait aucun mal à me suivre, dans la mesure

les suspects, les témoins -comme il se doit, avec toutes les précautions que nous avons prises, celles que votre commission a envisagées et celles que l'Assemblée nationale a votées, plutôt que de voir

Merci de me laisser respirer ... Pour le reste, ne pensez-vous pas qu'il soit utile que les Français sachent comment fonctionne une instruction, qui est le juge d'instruction, à quoi sert le greffier, à quoi sert l'avocat aux côtés du mis en examen ?

et vous la négligez, comme si ce que vous proposiez était l'alpha et l'oméga de la pédagogie sur ce qu'est la justice dans notre pays. Cela ne suffit pas

il est écrit : « Il est vrai qu'à ce jour l'impact de ces tournages, s'ils devaient se généraliser, n'est pas connu. » Et encore : « Les rapporteurs ont exprimé leurs doutes sur l'objectif réel et l'opérabilité d'un dispositif conçu avant toute chose pour être un instrument de communication du ministère de la justice, tout en reposant sur l'intervention de producteurs et diffuseurs tiers pour éviter d'avoir à faire supporter par le budget du ministère les frais de tournage et de diffusion. » Je continue de citer le rapport : « L'article 1 ne semble avoir fait l'objet d'aucune concertation avec les professionnels.

Cet amendement vise à étendre l'enregistrement de l'audition, au cours d'une enquête, à toutes les victimes de délits et de crimes sexuels, quel que soit leur âge. Actuellement, cette disposition n'est prévue que pour les victimes mineures. Nous proposons d'élargir cette possibilité à l'ensemble des victimes de violences sexuelles, que ces victimes soient mineures ou majeures. L'adoption de cet amendement permettrait d'éviter à une victime majeure d'avoir à relater à plusieurs reprises les violences sexuelles qu'elle a subies, lui épargnant l'effet traumatique d'une telle répétition.

a pour objet de limiter l'application des délais de trois et deux ans aux enquêtes sur les faits de corruption internationale

y compris dans le domaine économique et financier, m'apparaît de nature à améliorer l'efficacité de l'action de la justice et à accroître la sécurité juridique des personnes mises en cause, la question peut toutefois se poser de l'extension des exceptions prévues à l'heure actuelle dans la petite loi au seul domaine de la lutte contre la corruption internationale, compte tenu des spécificités propres à la conduite de l'action publique en ce domaine et de sa particulière sensibilité politique.

autant, quand une enquête préliminaire ne sera pas terminée dans les délais nouveaux que vous fixerez, alors on basculera automatiquement vers

sous une autre forme, en l'occurrence l'instruction. Je pense qu'il ne faut pas multiplier les exceptions ; nous risquons de nous y perdre et de faire perdre à ce texte

Le combat contre ces crimes et délits est une cause nationale. Les enquêtes peuvent parfois concerner des personnes étrangères, comme c'est le cas dans les trafics d'êtres humains.

Merci,

pour le bon fonctionnement de la société. Si j'étais un peu excessif, je dirais qu'une enquête préliminaire qui durerait trop longtemps résulterait soit d'une inertie anormale soit d'une forme de pathologie technique.

l'oral du concours a été supprimé, ce qui veut dire qu'on recrute des enquêteurs judiciaires, dont, je le rappelle, les responsabilités sont importantes, sans avoir pu tester leur personnalité, leur manière d'être. Monsieur le garde des sceaux,

que, s'il est un spécialiste des affaires financières, c'est bien le patron du parquet national financier, que nous avons consulté. Il a écrit à mes services, le 28 juin 2021,

réalisée dans le secret absolu, sans qu'à aucun moment la personne susceptible d'être renvoyée un jour à l'instruction ait la possibilité de s'exprimer. Je pense profondément que l'enquête préliminaire a été créée parce que le parquet a la lourde responsabilité de décider de transférer ou non devant un juge d'instruction.

de se défendre dès le départ ; cela permet sans aucun doute de gagner du temps, car des explications sont apportées, ce qui est strictement impossible dans l'enquête préliminaire. C'est la raison pour laquelle j'incite mes collègues à accepter l'idée que l'enquête préliminaire

L'étude d'impact du projet de loi souligne, à ce sujet, que, dans la plupart des pays européens, « parmi les droits les plus fréquemment conférés à la personne au cours de l'enquête figurent le droit d'accès au dossier, le plus souvent au cours de la garde à vue, et le droit de demander des actes d'enquête ou de participer à des actes d'enquête et d'être informé de ses droits. Cet amendement s'inscrit dans la lignée de la position de notre groupe : une justice plus efficace ne doit pas se faire au détriment des droits des justiciables. Le Gouvernement souhaitant raccourcir les délais de l'enquête préliminaire en alléguant l'amélioration parallèle des droits de la défense, en matière d'accès au dossier notamment, il ne trouvera, à notre avis, rien à redire à cet amendement, qui s'appuie d'ailleurs sur des travaux du Conseil national des barreaux

de la commission ? Cet amendement a passionné l'Assemblée nationale, qui ne l'a cependant pas retenu. Vous savez que les droits de la défense sont garantis au cours de la garde à vue, puisque l'avocat est présent et que la personne suspectée est informée de la qualification et de la date de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise. Surtout, elle est informée de son droit de garder le silence.

Il vise à bien préciser dans le texte que les dispositions relatives à l'ouverture de l'enquête préliminaire au contradictoire s'appliquent que l'intéressé soit soupçonné d'avoir commis une infraction en tant qu'auteur ou en tant que complice. monsieur le rapporteur.

au suspect et à son avocat dès le stade de la garde à vue ou de l'audition libre. Au regard du droit à un procès équitable, le droit d'accès au dossier pour le citoyen mis en cause dans le cas d'une enquête préliminaire apparaît en effet indispensable. L'étude d'impact du projet de loi souligne d'ailleurs, à cet égard, que, dans la plupart des pays européens, « parmi parmi les droits les plus fréquemment conférés à la personne au cours de l'enquête figurent le droit d'accès au dossier, le plus souvent au cours de la garde à vue, et le droit de demander des actes d'enquête ou de participer à des actes d'enquête et d'être informé de ses droits Le suspect et son avocat, avant la garde à vue ou l'audition libre, devraient donc pouvoir avoir accès au dossier de l'enquête, expurgé, bien évidemment, des éléments devant rester secrets dans l'attente de la fin de l'investigation en cours et ne pouvant être connus que des enquêteurs, afin que le suspect puisse avoir la meilleure connaissance possible, à ce stade de l'enquête, des charges et indices qui pèsent sur lui.

que nous avons accepté sans présenter aucun amendement, à savoir l'ouverture au contradictoire, qui intervient au bout d'un an. Nous pensons qu'il y a là un bon équilibre, si je puis dire, entre les positions qui ont été exprimées.

Oui, mes chers collègues, si l'on parle de la relation entre l'avocat et son client, ou entre l'avocat et les tiers. En revanche, ce secret professionnel n'est pas absolu lorsqu'il se confronte avec l'autorité régalienne, avec le pouvoir judiciaire, dans un cadre assez simple où deux principes constitutionnels s'entrecroisent.

Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le rapporteur : c'est incessible ; c'est insécable ; c'est inaliénable ; c'est indivisible ; c'est intouchable ; c'est sacré. C'est comme ça ! C'est l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui en dispose

ou d'assistance, bénéficie de ce secret. Ce secret s'entend comme un tout : il couvre toutes les matières du droit, dans tous les domaines d'activité de l'avocat, que l'on parle de consultation, de correspondance, d'entretien ou de défense.

L'introduction de cet alinéa en commission des lois induit une confusion délétère et dangereuse, nous semble-t-il, entre, d'une part, les pièces d'un justiciable, qui ne sont pas couvertes par le secret professionnel de l'avocat et sont donc saisissables dans le cadre des enquêtes pénales si cela est utile à la manifestation de la vérité, et, d'autre part, les consultations d'avocat, les correspondances entre avocat et client, ainsi que les factures adressées par l'avocat au client, qui sont couvertes par le secret et ne doivent en aucun cas pouvoir être saisies, sauf si elles recèlent la preuve de la participation de l'avocat à une infraction pénale. En outre, véritable sanctuaire pour l'exercice même de la profession d'avocat, le secret professionnel repose sur la garantie de deux droits fondamentaux : le droit de se confier à un avocat sans crainte que ces confidences soient un jour utilisées contre son consentement et servent et servent de fondement à une incrimination, corollaire du droit de ne pas s'auto-incriminer ; le droit de recueillir les consultations juridiques d'un avocat en toute matière sans crainte de voir un jour ces consultations utilisées contre soi. Plus largement, en portant atteinte à l'indivisibilité du secret professionnel des avocats, c'est la légitimité même de l'État de droit que l'on affaiblit, en ce que celle-ci repose, entre autres, sur le respect par les autorités publiques du secret professionnel de l'avocat en toute matière. Enfin, et surtout, si le présent projet de loi affiche pour ambition de rétablir la confiance, aujourd'hui dégradée, de nos concitoyens dans la justice, cette disposition va à rebours de l'esprit du texte en sapant précisément la confiance qu'ils peuvent avoir envers les avocats et la justice.

des droits fondamentaux, à la fois pour le client et pour l'avocat, qui est d'ailleurs protégée par le droit européen, en matière tant de défense que de conseil. Qui dit secret professionnel dit confidentialité, secret de l'échange entre un avocat et son client.

et de qualité, et donc d'une meilleure application de la règle de droit dans la société. La confiance est au coeur du secret professionnel. Elle est indispensable au bon fonctionnement de notre système judiciaire. Elle est d'ailleurs au fondement de ce texte, puisqu'il est justement question de restaurer la la confiance dans l'institution judiciaire. Je ne peux que saluer les dispositions de ce projet de loi qui renforcent la protection du secret professionnel de l'avocat. Il est pertinent que celui-ci soit étendu aux activités de conseil, afin de couvrir tout le champ

à raison de la nature des infractions lorsque l'avocat n'a pas participé à la commission des infractions poursuivies. Rappelons un point qui fait consensus : le secret professionnel est d'ores et déjà inopposable dans le cas où l'avocat est soupçonné de participer à la commission d'une infraction. Aussi, je crains que l'adoption de l'amendement de la commission n'ait pour effet de limiter le secret professionnel de l'avocat, ce qui ne peut se faire qu'au préjudice du justiciable et de la force de notre État de droit. Le secret professionnel de l'avocat doit être

avaient tranché dans le sens que vous indiquez, au regard de la primauté du droit européen, il n'y aurait pas matière à se réunir, car le droit français aurait été mis en conformité. la situation, aujourd'hui, n'est pas celle que vous avez décrite. Je passe très vite là-dessus : Cour de cassation, 24 novembre 2020,

illimitée- quand, je le rappelle, nous proposons simplement de l'étendre -, vous ne permettez pas à notre société de lutter correctement contre la corruption ou la fraude fiscale.

le plus sincère est que, dans le cadre de la navette parlementaire, on puisse enfin trouver, sur cette question, le meilleur des compromis.

J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'intervention de notre rapporteur, qui est un homme convaincu et de bonne foi. Depuis la loi de 1971, le monde a changé. le monde a changé. La mondialisation de l'économie, la rapidité des échanges d'informations et des flux internationaux, la multiplication des déplacements donnent à l'ordre économique international des capacités d'intervention qui sont extraordinaires et, en apparence, difficiles à contrôler. Mais il ne s'est pas rien passé entre 1971 et 2021.

l'expression d'un secret professionnel sans limite en faveur des avocats pour ce qui est des activités non liées à la défense, le Conseil constitutionnel nous rappellerait

donc qu'il nous faut rester détendus. Il vaut mieux que nous écrivions nous-mêmes, de la façon la plus soigneuse possible, la délimitation de ce secret professionnel en matière de conseil, plutôt que de devoir appliquer

de la société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur un défenseur, le catholique un confesseur, mais ni le médecin, ni l'avocat, ni le prêtre ne pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites n'étaient assurées d'un secret inviolable. » Je me mets à la place

Cela dit, je ne suis pas d'accord avec notre collègue Jean-Baptiste Blanc lorsqu'il affirme que le secret de l'avocat est absolu depuis 1971. Telle n'est pas la vérité

Le scrutin est clos.

vous avez d'ailleurs régulièrement dénoncées, à juste titre, lorsque vous étiez encore avocat. Par cet amendement, je vous propose que que les éléments collectés lors d'une surveillance téléphonique ou électronique ne puissent être utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles le juge des libertés et de la détention a autorisé Vous l'aurez compris, mes chers collègues, il s'agit de renforcer le secret professionnel entre le client et son avocat, sans lequel les droits de la défense ne peuvent être correctement assurés. Lorsqu'un client échange avec son avocat, avec son médecin, d'ailleurs, il lui confie ce qu'il a de plus cher : son honneur, sa santé, sa liberté, sa dignité. Si nous voulons garantir à tout citoyen l'absence d'ingérence des pouvoirs publics dans sa défense, nous devons préciser plus avant les contours du secret professionnel.

les dispositions dont nous venons de débattre.

La présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu est requise. Dans certains cas, la personne retenue sera sommée de fournir des renseignements, y compris auto-incriminants.

le déroulement des enquêtes ; à mon sens, ils perdent en partie de vue l'objectif de notre système judiciaire. La présomption d'innocence, chère à tous, est en effet garantie par les droits de la défense tout au long de la procédure. L'avocat est trop souvent perçu comme un élément perturbateur des enquêtes alors qu'il est un rouage essentiel de l'équilibre des procès.

-l'obligation pour les enquêteurs de rappeler à la partie qu'elle a le droit de se taire et, partant, de ne pas s'auto-incriminer. Cela

étant, nous regrettons l'alourdissement des sanctions prévues à cet article, alors que les condamnations en la matière sont aujourd'hui marginales. Une fois de plus, le Gouvernement semble afficher des objectifs contradictoires. Il réaffirme l'importance du secret de l'enquête,

légitimement les informations issues de cette enquête ou instruction. Par voie de conséquence, une telle absence de garantie pourrait entraver l'exercice des droits de la défense. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet article. Quel est l'avis de

sénateurs, cet amendement a pour objet de rétablir l'article 5 du présent texte, qui tend à favoriser le recours à l'assignation à résidence sous surveillance électronique en lieu et place de la détention provisoire. J'ai été un peu surpris de constater que votre commission des lois avait adopté un amendement de Mme Boyer de rétablir l'article 5 du présent texte, qui tend à favoriser le recours à l'assignation à résidence sous surveillance électronique en lieu et place de la détention provisoire.

-chaque fois qu'elle apparaîtra indispensable comme mesure de sûreté, notamment pour éviter de nouveaux faits ou à raison de nécessités de l'instruction. Il ne s'agit pas de remplacer la détention par la surveillance électronique mobile : nous voulons simplement que cette surveillance soit prononcée chaque fois que la détention peut être évitée. concerne le recours au bracelet anti-rapprochement en cas de violences au sein du couple, votre commission indique, dans son rapport, que ce dispositif connaît des difficultés et peine à être mis en oeuvre du fait d'un manque de bracelets disponibles. C'est totalement inexact ! Il est vrai Il est vrai que cette mesure nouvelle est appliquée de manière progressive par les juridictions ; mais en aucun cas les magistrats souhaitant y recourir ne voient leur action entravée faute de matériel.

d'une surveillance électronique ou d'un bracelet anti-rapprochement. Il rendait également obligatoire la saisine du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) avant la date de la seconde prolongation de la détention provisoire, lorsque l'intéressé encourt une peine d'emprisonnement de cinq ans ou moins.

La détention provisoire est aujourd'hui l'exception. Nous l'avons voulue comme telle. Elle ne devrait être prononcée que lorsqu'elle s'avère nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête. La percevoir comme le début d'une punition nuit totalement aux mis en cause. Corollaire de la présomption d'innocence,

que le sens de la détention et de la contrainte participe de la motivation de l'encadrement des décisions de prolongation de la détention provisoire, encadrement que cet amendement vise à rétablir.

Rappelons, à cet égard, que les rapporteurs n'avaient pas eux-mêmes déposé d'amendements sur cet article dont la suppression est intervenue via l'adoption d'un amendement dont ils n'étaient pas les auteurs. Il faut enfin rappeler que les dispositions de l'article 5 n'interdisent en rien de recourir à la détention provisoire chaque fois que celle-ci s'avérera nécessaire. Je demande donc à mon tour le rétablissement de cet article.

à quelque moment que ce soit de la procédure pénale, la motivation du choix d'enfermer une personne en regard d'une autre mesure pouvant être effectuée en milieu libre. Cette disposition préserve l'office du juge, mais impose une obligation de motivation circonstanciée de l'emprisonnement comme dernier recours, car le juge est tenu d'examiner les raisons de l'impossibilité de prononcer une mesure en milieu libre. Il est en effet grand temps de réfléchir à des logiques de décroissance carcérale et de penser l'organisation de l'administration pénitentiaire sous l'angle de la régulation

Nous devrions en tirer le bilan, sachant par ailleurs que de telles logiques sont déjà déployées dans certains centres pénitentiaires, comme nous l'apprend la section française de l'Observatoire international des prisons. Quant à l'amendement il s'agit d'une recommandation du réseau d'associations Citoyens et Justice -, il vise à mentionner spécifiquement dans le texte la possibilité de soumettre le prévenu à des obligations socio-éducatives afin que soit engagé un travail sur ces problématiques- mobilisation autour du soin, d'une prise en charge psychologique, etc. etc. La structure désignée pour ce suivi produira obligatoirement un rapport avant l'audience de jugement, comportant des informations relatives à la situation du prévenu, aux actions engagées avec lui, à son adhésion à certaines mesures, à la faisabilité de certaines peines alternatives ou encore à sa capacité à respecter des obligations. Ces éléments se révèlent particulièrement utiles au tribunal dans son appréhension fine du prévenu, concernant tant la propension de ce dernier des mesures contraignantes que son engagement dans un travail visant à prévenir la récidive. Quel

Le code de procédure pénale prévoit déjà les garanties que vous souhaitez. Il le fait simplement dans une rédaction un peu différente : « Les mesures de contrainte dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. » Nous voyons bien, dans cette rédaction,

cet amendement revêt à mes yeux une importance toute particulière. Ils étaient deux. Ils ont été condamnés à trois reprises pour le meurtre d'un garde-chasse à la suite d'aveux qui leur avaient été extorqués

et ont été graciés par le président René Coty, mais n'ont jamais pu obtenir la révision de leur condamnation en dépit des six demandes qu'ils ont présentées. Ils sont morts à présent,

et pour que, même à titre posthume, l'injustice qui leur a été faite soit réparée. Je parle, bien sûr, de Mis et Thiennot. J'ai, comme vous sans doute, le souvenir

acharné contre une justice qui ne voulait pas dire qu'elle s'était trompée. La justice a dit à de nombreuses reprises la réalité des tortures mais elle a ajouté, suivant les textes de l'époque- ils ont été modifiés depuis -, que, puisque cette torture était connue lors du procès, elle ne constituait pas un élément nouveau susceptible de conduire à une révision.

pour des raisons de recevabilité et parce que nous n'y étions pas préparés, la mort dans l'âme, j'ai émis un avis défavorable.

l'Indre. Comme vous l'avez rappelé, ce drame s'est déroulé dans ce département, où deux innocents ont été condamnés après avoir été torturés pendant plus d'une semaine. MM. les députés Nicolas Forissier, qui ne pouvait pas être en séance, et François Jolivet ont déposé des amendements à ce sujet.

qui raccourcit, non plus la garde à vue- c'est chose faite, et heureusement, depuis longtemps -, mais la durée de l'enquête préliminaire, qui s'appelait, sous l'empire du code d'instruction criminelle, l'enquête officieuse.